En 2020, 2,17 millions d'heures ont été indemnisées pour un montant de 27,1 millions d'euros. Une partie de cette indemnisation s'est faite sur la base du volontariat, une autre de façon obligatoire en fin d'année, pour les agents ayant un solde d'heures supplémentaires supérieur à 500 heures.

que les conditions de travail qui leur sont proposées ne sont pas satisfaisantes, alors il faut faire un effort budgétaire, afin que ces heures supplémentaires leur soient payées. À un moment, il faut choisir

ou de vol en cas de mauvais temps. Ils ne garantissent pas pleinement la sécurité des victimes. Tous ces éléments ouvrent une faille dans la promesse républicaine. Il s'agit non pas de demander les mêmes moyens et les mêmes infrastructures que dans les métropoles- le prisme de l'égalité n'est ici pas le bon -, mais bien de réclamer l'équité. Les ruraux, quel que soit leur lieu d'habitation, en Lozère ou ailleurs, ne sont pas des sous-citoyens.

trente-quatre hélicoptères de la sécurité civile ne suffisent pas à couvrir l'ensemble du territoire et leur vieillissement peut provoquer de longues immobilisations pour maintenance, même si leur taux de disponibilité reste très élevé, de l'ordre de 95 %. La répartition des hélicoptères de secours sur notre territoire n'est pas satisfaisante, mais je ne suis pas certain que l'adoption de cet amendement résolve ce problème, pour deux raisons.

On sait aussi que leur implantation est parfois redondante avec celle des hélicoptères de la sécurité civile. Il faudrait donc que les ministères de l'intérieur et de la santé s'entendent sur une stratégie nationale et arrivent enfin à une flotte bleu-blanc-rouge qui garantisse un meilleur maillage du territoire. D'autre part, le ministère de l'intérieur a déjà entamé le renouvellement de sa flotte d'hélicoptères. Ainsi, 32 millions d'euros ont déjà été engagés en 2020 pour commander deux nouveaux hélicoptères, avec une livraison programmée pour Cette commande prévoit en outre deux appareils supplémentaires en option. Le ministère étudie enfin la possibilité d'acquérir prochainement deux hélicoptères de type lourd, d'un modèle plus performant et multi-rôle.

Nous connaissons, depuis quelques années, un accroissement sensible du nombre de personnels dans la police : c'est une bonne chose. Néanmoins, la formation doit

qu'un grand nombre de policiers n'ont même pas la possibilité de faire leur entraînement de tir annuel :

Nous saluons, évidemment, cette décision qui revient progressivement sur les milliers de suppressions de postes intervenues au cours du mandat de Nicolas Sarkozy. Il va sans dire qu'une présence accrue des gardiens de la paix sur le terrain devrait avoir un impact positif sur les chiffres de la criminalité et de la délinquance. Elle devrait également faciliter le quotidien des policiers surmenés, car en sous-effectifs. Cependant, force est de constater que l'emploi de ces nouvelles recrues ne s'est, hélas, pas accompagné d'une hausse des moyens alloués à leur formation. Cette situation est extrêmement problématique, d'autant plus que nous constatons, ces dernières années, une multiplication des faits de violence perpétrés par certains éléments des forces de l'ordre. Un devoir d'exemplarité doit être de mise pour chacun de nos fonctionnaires de police, une meilleure formation de ceux-ci ne pouvant qu'avoir un effet bénéfique sur leur comportement. En effet, une police mieux formée est une police sensibilisée qui enregistre les plaintes de manière adéquate, qui applique les consignes de la préfecture avec discernement et qui noue des liens sociaux courtois avec les concitoyens. Somme toute, une police mieux formée est une police qui protège mieux, car elle est à l'écoute des besoins de sa population. Alors que les tensions sont de plus en plus vives au sein de notre société, il est grand temps que notre police républicaine bénéficie de la formation qu'elle mérite. Il y va de notre sûreté à tous, comme de la sienne. Le présent amendement vise ainsi à renforcer, à hauteur de 20 millions d'euros, le programme 176, « Police nationale », afin de financer la formation des nouvelles recrues de l'institution policière. L'amendement

étant à la charge des collectivités territoriales. L'État ne participe qu'à hauteur de 950 millions d'euros, dont 520 millions issus du programme 161, « Sécurité civile ». Cela représente seulement 7 % de l'intégralité des dépenses en la matière. Pendant la crise du covid-19, les acteurs de la sécurité civile n'ont, pourtant, pas ménagé leurs efforts : les sapeurs-pompiers des

Alors que les catastrophes sanitaires et environnementales pourraient se multiplier dans les années à venir en raison du réchauffement climatique, il est nécessaire que l'effort financier engendré par les dépenses de sécurité civile soit mieux réparti entre les localités et l'échelon

», en particulier son action n° 13, Soutien aux acteurs de la sécurité civile. Quel

dans le budget et qu'il serait superflu de les augmenter, tant que nous n'avons pas les formateurs et que la décision inverse de celle qui a été prise par le passé n'est pas

puisque, par définition, l'exercice auquel nous nous livrons nous impose de gager nos amendements. Or je note que le Gouvernement ne lève pas le gage ... Soit nous considérons qu'il ne faut rien changer, et dans ce cas-là, à part le plaisir de partager une séance dans l'hémicycle, je ne sais pas ce que nous faisons là ; soit nous prenons nos responsabilités. On ne peut pas, à longueur d'interviews, de papiers et de déclarations officielles du ministre de l'intérieur, y compris devant la commission des lois du Sénat, dire que la formation est un problème,

Il en découle, aujourd'hui, des tensions indéniables entre les forces de l'ordre et nos concitoyens. En effet, la police nationale est mise en cause en raison des violences disproportionnées de certains CRS à l'encontre de manifestants lors des récents mouvements sociaux.

aurait également critiqué l'accroissement des contrôles au faciès sur certaines catégories de population, ce qui est une discrimination, selon le Défenseur des droits. Après les exactions commises, le soir du 23 novembre, par les forces de l'ordre lors de l'évacuation d'un camp de migrants place de la République, il est nécessaire que de nouveaux garde-fous soient mis en place. en place. Il s'agit de limiter les pratiques policières au respect de la stricte légalité et, ainsi, de sanctuariser la sécurité de nos concitoyens. Il est vital, aujourd'hui, de renouer un dialogue sain entre l'institution policière et notre société. Pour ce faire, de nouvelles pratiques peuvent être expérimentées. Le présent amendement a pour objet de financer, à hauteur de 10 millions d'euros, la généralisation de l'usage des caméras-piétons.

des propositions de loi pour lutter contre le contrôle au faciès. Nous sommes convaincus que de tels dispositifs seraient susceptibles de garantir des pratiques plus vertueuses de nos policiers ainsi qu'une plus grande transparence de leurs actions. Ces outils peuvent être la clé de la confiance retrouvée entre les Français et leur police républicaine. L'amendement

de la police nationale, il est toujours très mesuré. Il a déclaré récemment : « Le matériel acheté par le ministère est totalement inefficace. Aujourd'hui, la caméra est tellement bas de gamme qu'il faudrait partir avec quatre batteries pour tenir une vacation entière. Il faut un budget conséquent pour acheter du matériel de bon niveau. »

qu'elle est discriminée dans la façon dont elle est contrôlée. Je me fie aux chiffres établis par le Défenseur des droits sur le coefficient multiplicateur des contrôles à l'égard d'un certain nombre de populations jeunes et d'apparence

que défendre les droits et les libertés ou manifester n'est pas incompatible avec une exigence de soutien aux forces de police et de sécurité dans notre pays. pays. Je sais bien que certains ici ne manifestent ni pour soutenir les policiers ni pour défendre celles et ceux qui revendiquent leurs droits et leurs libertés dans ce pays. Frappés

est peut-être aussi le résultat de décisions prises voilà quelques années. Dès lors, mes chers collègues, ne méprisez pas les gens qui manifestent dans la rue pour soutenir les revendications des salariés et du peuple de France sur quelque question que ce soit

ce sont bien nos forces de sécurité de façon générale qui en paient les conséquences. Je voulais profiter de ce débat pour le dire avec solennité.

a aussi une mission d'enquête, lorsque le parquet ou un juge d'instruction décide de lui confier des investigations dans le cadre d'une enquête en cours.

très peu d'éléments budgétaires ont été transmis par le Gouvernement dans sa présentation du programme 176, « Police nationale », de la mission « Sécurités » du PLF pour 2021. Nous proposons

Je prendrai position

aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM). La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a institué des avances remboursables en faveur des AOM. Le dispositif prévu intègre le versement mobilité dans le panier des recettes fiscales prises en compte pour le calcul de la compensation financière. Toutefois, pour certains acteurs du transport public, la globalisation des recettes fiscales du budget général et des budgets annexes a pour effet de diluer le problème spécifique aux transports. Elle pénalise notamment les AOM organisées en EPCI à fiscalité propre, alors que les syndicats mixtes de transport, par exemple, verront leurs pertes de recettes fiscales compensées- et tant mieux pour eux. Cet amendement vise donc à mettre fin à une forme d'inégalité de traitement en prévoyant un abondement de 500 millions d'euros. Quel est

en installant notamment des radars " leurres ", mais également en augmentant le nombre de radars autonomes déplaçables et en augmentant l'utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés en confiant leur conduite à des prestataires La France dispose d'un réseau routier étendu, longtemps considéré comme exceptionnel, et qui continue de se développer. Ce réseau est un atout formidable pour la mobilité dans nos territoires, à condition d'être bien entretenu.

la relance passe par la capacité des conducteurs à circuler sur des routes en bon état. Il s'agit de créer un contexte qui favorise les déplacements, notamment professionnels, en réduisant le risque d'accident dû à l'infrastructure. Il importe donc d'affecter une part suffisante des investissements pour 2021 à cette priorité. C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à réduire les crédits affectés à la modernisation et au développement de nouveaux radars de 57,55 millions d'euros et à les réaffecter à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières, afin de permettre aux collectivités de financer l'aménagement des zones accidentogènes et de mieux entretenir

754 pour les collectivités territoriales et 278 millions à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf). Si votre amendement était adopté, il n'y aurait plus aucun investissement dans les nouveaux radars

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Richelieu disait que « la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire ». Sur ces questions d'immigration, d'asile, d'intégration qui remettent en cause

ces évacuations qui se répètent sans cesse, et par l'agitation politique organisée par des associations qui participent à la chaîne de l'exploitation de cette tragédie humaine Ce malaise sur la question migratoire et le reste, l'asile et l'intégration, prend racine dans l'impuissance de l'État à prendre à bras-le-corps « sans tabou ni angle mort » ces sujets qui relèvent au premier chef de la souveraineté nationale. N'est-il pas urgent, au titre de sa mission

Nous ne le savons pas, car l'État lui-même ignore combien d'étrangers en situation irrégulière se trouvent sur le territoire national. Le rapport d'information déposé en 2018 par nos collègues députés Kokouendo et Cornut-Gentille

Les notions d'immigration, d'asile et d'intégration obligent à se poser les questions essentielles de la souveraineté, de l'intérêt national et de la cohésion de la société.

Au regard de l'état du monde et des différences de niveau de vie, la France offre une qualité de vie rare- santé gratuite, éducation, logement. Il constate que la France n'aboutit pas à des résultats satisfaisants en matière d'intégration. Nous devons penser une politique globale et une stratégie qui ne soit pas l'apanage d'un seul ministère et recentrer le droit d'asile sur un petit nombre de véritables réfugiés, faute de quoi il mourra. En matière de regroupement familial, nous sommes loin des critères allemands, hollandais ou autres. En matière de soins, nous sommes le seul pays, avec la Belgique, à délivrer un titre de séjour pour soins à celui qui arrive jusqu'à nous dès lors que la prise en charge, dans son pays d'origine, n'est pas effectivement accessible. En cette période de covid, les Français doivent savoir que nous prenons en charge la santé des sans-papiers, des clandestins, au-delà de l'urgence. La norme en Europe est de limiter la prise en charge aux soins d'urgence, dès lors que le pronostic vital est engagé. Nos centres d'accueil sont beaucoup moins sommaires que ceux de la plupart des pays d'Europe. Il est certain que ceux qui sont déboutés de l'asile bénéficient ici de plus de prise en charge que dans la plupart des pays européens. C'est pour cela, du reste, que ceux qui sont déboutés du droit d'asile, les « dublinés », traversent les Alpes, les Pyrénées ou le Rhin. Depuis 1980, une trentaine de réformes de la législation relative aux étrangers a rendu d'une complexité extrême un droit qui n'a pas été conçu globalement, mais par sédimentation. Le résultat est un carcan juridique, juridictionnel, conventionnel et constitutionnel. Le pouvoir démocratique a été complètement dépossédé de sa capacité de décision. Le syndicat de la juridiction administrative (SJA) souligne que le droit de l'immigration souffre d'une illisibilité de la politique d'accueil et de séjour des étrangers. Les magistrats s'interrogent sur le sens de leur travail,

Des noyades en Méditerranée aux évacuations des camps d'infortune, en passant par l'exploitation des migrants et l'assassinat de Samuel Paty ou des malheureux chrétiens de Nice, il est vraiment temps que cela change. Madame la ministre, le voulez-vous vraiment ?

Je dois à la vérité de dire que ce budget a été régulièrement abondé, depuis plusieurs années, par le Gouvernement : pour ce qui concerne l'immigration régulière, c'est l'intégration qui a été favorisée ; pour ce qui est du droit d'asile, dont notre collègue Philippe Bonnecarrère parlera sans doute plus avant,

encore 25 % de ceux qui sont arrivés en France et qui bénéficiaient, dans le cadre d'une immigration régulière, d'une formation linguistique, ne sont pas parvenus à atteindre le niveau de langue minimal requis pour s'intégrer dans un pays.

l'aide médicale de l'État, seule façon de mesurer l'immigration irrégulière, est en augmentation de plus de 5 %. C'est terrible ! La réalité est que nous subirons toujours cette pression migratoire, si nous n'essayons pas de la contrôler. Or nous n'essayons pas véritablement. J'en donnerai deux exemples : en 2018,

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'année qui se termine fut pleine de bouleversements. La pandémie a perturbé le fonctionnement de très nombreux pays, dont la France. La lutte contre le virus a rendu crucial le contrôle des flux transitant entre les pays, mais également en leur sein même. Cette diminution de la circulation des personnes a évidemment eu de grandes conséquences sur la mission « Immigration, asile et intégration » que nous examinons aujourd'hui. aujourd'hui. L'immigration reste un sujet sensible pour bon nombre de nos concitoyens. D'après un sondage IFOP de janvier dernier, près de 80 % d'entre eux considèrent qu'il faut passer d'une immigration subie à une immigration choisie. L'immigration est une chance, à condition que la France conserve la maîtrise des flux. La lutte contre l'immigration irrégulière doit être une priorité, madame la ministre, car elle mine notre politique migratoire. Comme bien d'autres de nos collègues, les membres du groupe Les Indépendants sont particulièrement préoccupés de voir que les obligations de quitter le territoire ne sont que trop faiblement exécutées. Voilà plus de dix ans que leur taux d'exécution n'a jamais dépassé les 25 %. Comment accepter que la grande majorité des décisions judiciaires en la matière restent dénuées d'effet ? Quel message est ainsi envoyé aux réseaux ? et à l'intégration des immigrés en situation régulière., c'est l'ensemble de notre société qui en pâtit. Nous savons que vous y travaillez, madame la ministre. Nous avons suivi avec attention vos démarches pour obtenir de meilleurs résultats sur la délivrance de laissez-passer consulaires, notamment Il faut poursuivre ces efforts pour parvenir à exécuter les obligations de quitter le territoire et, dans le même temps, concentrer nos efforts au profit de ceux que nous accueillons. Le droit d'asile est l'une des traductions de l'engagement de la France en faveur de la liberté. Réduire fortement le délai de traitement des demandes est à ce titre un objectif capital. Et nous avons tous à y gagner. Il faudra cependant se donner les moyens de l'atteindre. Les effectifs de l'Ofpra ne stagnent pas, mais se réduisent légèrement. Dans ces conditions, comment réussir à passer d'un délai d'examen de 112 jours, prévu pour 2021, à un délai de 60 jours en 2023 ? À cet égard, l'augmentation des crédits risque de ne pas être suffisante cette année. Nous notons que le plan de relance prévoit des investissements pour améliorer l'hébergement des demandeurs d'asile, mais le recours au plan n'est pas une solution soutenable. Nous devrons investir davantage dans la politique de l'immigration et de l'intégration si nous voulons parvenir à maîtriser pleinement la situation. Je veux rappeler aussi que la prise en charge des mineurs isolés coûte environ 2 milliards d'euros aux départements chaque année. Dans la mesure où seul l'État dispose du contrôle des frontières de notre pays, il nous semble que les dépenses engagées par les départements pour cette prise en charge devraient au minimum être compensées par l'État. Rien ne justifie que les départements en supportent le coût. Pour réussir le défi de l'intégration, notre pays doit assumer pleinement d'exercer un contrôle strict sur sa politique migratoire et se donner les moyens d'y parvenir. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la covid-19 a engendré de graves dysfonctionnements au sein de l'administration française, démontrant au passage la défaillance criante des pouvoirs publics à l'égard des personnes migrantes, notamment dans les centres de rétention administrative (CRA), devenus de véritables clusters.

Ce budget n'évite pas certains écueils des années précédentes. Il en est notamment ainsi du traitement de la lutte contre l'immigration irrégulière, dont le budget augmente de 16 % en crédits de paiement, soit une hausse de 68,1 68,1 % depuis 2017. Il est grand temps qu'un virage humaniste soit de mise sur cette thématique. En ce sens, nous approuvons la création de 6 000 places cette année dans les centres d'hébergement d'urgence pour migrants, ainsi que la légère hausse du budget pour les dispositifs d'intégration et d'accueil sur le sol français. Ces signes sont encourageants, quoique timorés. Heureusement que les associations sont là pour nourrir les migrants qui dorment encore dans la rue. Nous ne pouvons pas nous permettre d'appréhender la question de l'immigration et de l'accueil sous le seul prisme de la comptabilité budgétaire. Ce qui manque au Gouvernement, c'est une vision globale et surtout de long terme. Globale, tout d'abord, car cela fait des années que nous sommes incapables de réformer, avec les autres pays européens, le règlement de Dublin qui met les personnes migrantes dans des situations de précarité et de détresse indignes des valeurs défendues par l'Union européenne. Sur le long terme, ensuite, parce que les moyens accordés à l'Ofpra ne sont pas suffisamment ambitieux pour affronter les flux migratoires qu'engendreront les dérèglements climatiques des décennies à venir. Selon certains experts, d'ici à 2050, près de 1,5 milliard de réfugiés environnementaux pourraient tenter de rejoindre l'Europe. Madame la ministre, nous saluons les timides efforts que comprend ce PLF pour 2021, notamment en matière d'accès au droit d'asile et à l'intégration, mais aussi en termes de création de places d'hébergement pour les exilés. Cependant, une fois encore, le budget de cette mission fait la part belle à la lutte contre l'immigration irrégulière. Par ailleurs, les faits de violences policières sur des migrants, perpétrés le 23 novembre dernier, démontrent que l'approche gouvernementale en matière d'immigration reste répressive. Ainsi, les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires voteront contre le budget de la mission « Immigration, asile et intégration ». La parole

Il traduit les dispositions de la loi du 10 septembre 2018, s'inscrit dans la dynamique impulsée par le comité interministériel du 5 juin 2018 et vise deux grands objectifs : mieux accueillir les demandeurs d'asile et les étrangers en situation régulière et lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Pour atteindre le premier objectif, le budget prévoit la structuration et la hausse du parc d'hébergement des demandeurs d'asile, qui sera doté de 6 000 places supplémentaires. Les campements indignes de migrants que l'on voit fleurir sur notre territoire nous montrent à quel point il est nécessaire de poursuivre nos efforts pour améliorer notre dispositif d'accueil. À cet égard, je sais M. le ministre de l'intérieur choqué par les violences inacceptables survenues place de la République lors de l'évacuation du campement qui s'y était installé. Je ne doute pas qu'il saura faire la lumière sur ce qui s'est passé et prendre les décisions qui s'imposent. Par ailleurs, il me semble important de rappeler que ces crédits sont examinés dans un contexte sanitaire exceptionnel, qui, compte tenu des restrictions de déplacement depuis mars dernier, a bien évidemment eu un impact sur le nombre de demandes d'asile qui ont été présentées cette année. C'est la raison pour laquelle je tiens à saluer le fait que le Gouvernement en ait tenu compte, en retenant, pour évaluer la demande d'asile en 2021, les chiffres de 2019. L'augmentation significative de l'allocation pour demandeur d'asile est, à ce titre, à souligner. Ce budget permettra également de poursuivre l'effort de maîtrise des délais de traitement des demandes d'asile, en consolidant les moyens supplémentaires accordés à l'Ofpra. Concernant le second objectif que représente la lutte contre l'immigration clandestine, les crédits sont consacrés pour une large part à l'investissement immobilier des CRA et à l'éloignement de ceux qui se maintiendraient illégalement sur le territoire. Je finirais mon intervention, une fois n'est pas coutume, en évoquant la situation à Mayotte, alors qu'un nouveau drame a eu lieu voilà deux mois, entraînant la mort de dix migrants, dont un enfant, tous venus des Comores. Vous le savez, sur ce territoire, la pression migratoire est telle qu'elle compromet absolument tout développement. Elle engendre paralysie des services et politiques publiques, crée des conflits entre communautés, et une montée mécanique de la délinquance. Le nombre de mineurs isolés et non accompagnés dépasse les chiffres les plus alarmants rencontrés en métropole. Comment Mayotte, dont chacun connaît la problématique migratoire spécifique, s'insère-t-elle dans la stratégie de la mission pour l'année 2021 ? au retour (DPAR) et des CRA se déclineront-elles au sein de ce département et, plus globalement, dans les territoires ultramarins ? Le 26 août dernier, j'avais adressé au Premier ministre un courrier faisant état des difficultés rencontrées à Mayotte en matière d'immigration et des conséquences de cette dernière sur les politiques publiques. J'y avais proposé des mesures concrètes. M. le ministre de l'intérieur en avait également été destinataire, et je lui sais gré de m'en avoir accusé réception. Pouvez-vous me dire, madame la ministre, si certaines d'entre elles ou même la totalité - j'ose être optimiste ! - ont d'ores et déjà été prises en considération, bien évidemment en lien avec M. le ministre des outre-mer ? En conclusion, et pour revenir spécifiquement aux crédits de la mission, nous observons que le Gouvernement maintient les efforts engagés depuis le début de cette législature pour répondre à une politique migratoire juste. C'est la raison pour laquelle le groupe RDPI votera les crédits de cette mission.

étrangers, réfugiés, migrants, exilés, demandeurs d'asile, ou encore clandestins et sans-papiers. Mais, au-delà des mots, nous parlons d'abord de femmes, d'hommes et d'enfants, qui méritent que notre nation leur réponde par une politique claire, digne et à la hauteur des valeurs républicaines et humanistes que nous défendons. Aussi, le budget dont nous discutons les crédits est une chance pour le débat démocratique : si ses enjeux sont actuels, ils concernent aussi le long terme pour notre pays, compte tenu de l'importance qui s'attache à la définition d'une politique d'intégration acceptable. À l'heure où l'Union européenne entend donner un nouveau cadre à la politique migratoire, nous voulons saluer l'effort fourni au travers de la hausse des crédits. La stabilité de ceux qui sont dévolus au logement ou à l'emploi des réfugiés ayant besoin d'un accompagnement spécifique reste un signal positif, alors que le contexte budgétaire est, nous le savons, très dégradé par ailleurs. Toutefois, quelques inquiétudes demeurent. Je pense d'abord aux administrations ayant la charge de l'accueil des ressortissants étrangers qui arrivent sur notre territoire. Alors que le nombre de demandeurs connaît une hausse continue, l'OFII et l'Ofpra doivent pouvoir exercer leur mission efficacement et dans des conditions respectant la dignité de leurs usagers. Si, s'agissant de l'Ofpra, nous observons avec satisfaction que son financement est en hausse, la situation de l'OFII est plus préoccupante, puisque ses subventions diminuent. Or, outre les difficultés qu'il pouvait connaître jusqu'alors, l'Office souffre de la pandémie et peine à répondre aux sollicitations des demandeurs d'asile et des réfugiés. La baisse de ses moyens dans ce contexte complexe nous étonne autant qu'elle nous inquiète. S'agissant par ailleurs de la gestion de l'immigration irrégulière, je ne suis pas la première à attirer votre attention, madame la ministre, sur la situation préoccupante des centres de rétention administrative, qui suscitent régulièrement la condamnation de l'État et des injonctions du juge administratif. La crise du covid-19 nous force à traiter le problème de la promiscuité dans ces centres, d'autant que la fermeture des frontières place ceux qui y sont retenus dans un état d'attente préoccupant. Le Défenseur des droits avait alerté très tôt, dès le mois de mars, sur cette question. S'agissant ensuite de l'immigration régulière, qui est elle aussi en hausse continue, se pose mécaniquement la question de l'intégration des nouveaux arrivants et des moyens qui y sont alloués. Nous le disions déjà lors de nos discussions sur la loi du 10 décembre 2018, aucune intégration sur le territoire de la République ne pourra se faire si l'on ne veille pas à ce que les personnes présentes sur ce territoire parlent français, connaissent la société française et en respectent les règles. Il faut donc que les crédits alloués le permettent. De ce point de vue, je crains que ce budget n'atteigne pas ces objectifs, pourtant fondamentaux pour mon groupe, qui est très attaché à défendre une République unie et apaisée. Enfin, tous nos efforts resteront vains s'ils ne trouvent pas d'écho au niveau de l'Union européenne. Alors que la présidente de la Commission européenne a mis en oeuvre depuis le mois de septembre une réforme profonde de la politique migratoire, celle-ci suscite de nombreux débats, voire l'opposition de certains États membres, au risque de mettre à mal la solidarité européenne. Il est crucial que la France s'engage pour une juste répartition des efforts d'accueil et d'intégration, toujours dans la dignité, mais aussi sans remettre en cause notre conception universaliste de la société autour des valeurs de la République. Ces remarques faites, mes collègues du groupe du RDSE et moi-même ne nous opposerons pas au budget qui nous est proposé.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que la majorité sénatoriale s'inquiète de « la multiplication des demandes d'asile obéissant à des motifs socio-économiques plutôt qu'à des motifs politiques et du faible nombre d'éloignements auquel il est procédé », nous nous nous préoccupons, pour notre part, du manquement grave de notre pays à ses obligations en matière d'asile, notamment en matière d'accueil, et de la politique d'enfermement des migrants, opérée également à l'encontre des enfants. Aussi, je vous le dis d'emblée, si nous nous opposons vertement aux crédits de cette mission « Immigration, asile et intégration », nos motifs sont diamétralement opposés à ceux des rapporteurs et de la commission des lois.

Dans la droite ligne des réformes précédentes, cette loi a accentué la mise sous contrôle des demandeurs d'asile et multiplié les obstacles et les contrôles entravant, de fait, l'accès des étrangers à leurs droits fondamentaux. Je ne peux aborder l'ensemble de la problématique, mais je voudrais aujourd'hui insister sur la question de l'hébergement des demandeurs d'asile et sur celle de l'enfermement des migrants. Après 66 évacuations de campements depuis 2015 à Paris, l'évacuation brutale, place de la République, la semaine dernière, a mis en relief les dysfonctionnements de la politique d'asile en France : près de la moitié des demandeurs d'asile ne sont pas pris en charge. Telle est la réalité. Malgré les créations de places de ces dernières années, le dispositif national d'accueil pour demandeurs d'asile reste marqué par un important sous-dimensionnement. En octobre, selon l'OFII, 147 400 demandeurs d'asile ont reçu une allocation mensuelle, alors que la capacité d'accueil au sein du dispositif national d'accueil s'élève à 81 81 119 places. Ainsi, plus de 66 000 demandeurs d'asile seraient privés de prise en charge. Cela va sans dire, les 4 500 places supplémentaires prévues dans ce budget ne permettront pas de rattraper le retard. À cela s'ajoute la crise sanitaire en cours, qui, d'une part, fausse les chiffres, les prévisions, et donc le budget pour 2021, et, d'autre part, dégrade davantage les conditions sanitaires des campements de fortune rendus encore plus insalubres. Il en est de même dans les centres de rétention administrative et dans les zones d'attente : la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et l'Observatoire de l'enfermement des étrangers ont demandé dans ce contexte que soient libérés immédiatement les retenus. En vain De nombreuses associations, dont Médecins du monde et Amnesty International, dénoncent la banalisation de la privation de liberté des personnes étrangères. Cette politique « punitive » du Gouvernement envers les étrangers détenus dans les centres de rétention administrative entraîne des tensions et des drames : grève de la faim, émeutes, automutilation, tentatives de suicide ... Pourtant, le Gouvernement s'entête en augmentant encore avec ce budget le nombre de places prévues dans les 21 CRA du pays. Ainsi 480 places supplémentaires sont-elles budgétisées. Dans ces CRA, on continuera de compter des enfants, car le Gouvernement et sa majorité persistent également dans leur refus d'interdire l'enfermement des enfants, en dépit des condamnations multiples de la Cour En 2019, 136 familles, dont 279 enfants, ont été enfermées en rétention en métropole, et plus de 3 000 à Mayotte ! Le drame humain qui se joue dans l'échec de notre politique migratoire n'est pas digne de nos grands principes républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en réaction à ce que j'ai entendu de la part de certains de nos rapporteurs, je souhaiterais d'abord rappeler certains chiffres tirés des données d'Eurostat. Concernant les délivrances des premiers titres de séjour, nous sommes au vingt-troisième rang en Europe, proportionnellement au nombre de nos habitants. En chiffres bruts, avec 274 000 premiers titres de séjour en France, nous sommes derrière la Pologne, qui en délivre 724 000, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Un tiers des titres que nous délivrons sont destinés à des étudiants et un sixième à des familles de Français.

Contrairement à nos partenaires et singulièrement à l'Allemagne, nous n'avons pas eu d'à-coups brutaux, mais une progression régulière, je dirai même prévisible, pour atteindre le chiffre de 120 000 primo-demandeurs en 2019.

en juillet, pour traitement dégradant de demandeurs d'asile. Au printemps, tirant prétexte de la crise sanitaire, le Gouvernement tentait, par ordonnance, d'élargir la possibilité de juge unique à la CNDA. Heureusement, le Conseil d'État veillait ! Pendant ce temps, les centres de rétention n'ont pas été correctement adaptés à la crise sanitaire.

Ces risques et ces humiliations, parfois pendant plus de deux mois, pour moins de 40 % d'éloignements, c'est indigne ! Madame la ministre, avant, il y avait des queues devant les préfectures. C'était insupportable, mais il suffisait d'attendre. Aujourd'hui, c'est la justice qu'il faut saisir pour avoir un rendez-vous en préfecture. préfecture de nouvelle génération rime avec préfecture virtuelle, tant la prise de rendez-vous en ligne est défectueuse. Comment enregistrer une demande d'asile ? Comment renouveler une carte de séjour ? Comment demander une autorisation exceptionnelle de séjour quand la crise sanitaire vous empêche de rentrer chez vous ? ? Ces remarques pourraient aussi concerner la plateforme d'appel de l'OFII. Comment, madame la ministre, construire l'image de la République avec ce type de défaillances ? Après des années à nous être acharnés à réduire les délais d'instruction des demandes d'asiles, n'est-il pas temps de constater qu'il existe un temps minimum incompressible pour l'étude des dossiers et qu'il serait utile qu'il soit consacré à la préparation de l'éventuelle intégration de la personne ? Je pense à l'apprentissage de la langue, à la formation, au droit au travail. Sans préparation à l'intégration, comment s'étonner que plus de 60 % des places de CADA soient occupées par des personnes ayant le statut de réfugié, qui ne peuvent aller ailleurs, faute d'avoir commencé un parcours d'intégration pour devenir autonomes ?

cette année. Je formulerai quelques remarques liées à l'actualité. Il est essentiel que l'Ofpra soit présent lors des audiences à la CNDA, lorsque sa décision initiale de refus de protection s'appuie sur une alerte sécuritaire. Cela doit être pris en compte de manière systématique, dans le respect du contradictoire, lorsque la juridiction de la CNDA prend ses décisions. décisions. Plutôt que de mettre en réadmission « Dublin » vers l'Italie des personnes en besoin de protection, il est grand temps que nous marquions notre solidarité totale avec ce pays. C'est une question d'humanité, d'efficacité et de crédibilité dans les négociations actuelles sur le prochain paquet Asile. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, un rapport de l'Assemblée nationale rappelle le coût moyen d'une expulsion, à savoir 15 000 euros, soit une année de SMIC net. Dès lors, pourquoi pourquoi s'acharner à développer les départs forcés, alors que les départs volontaires sont moins coûteux, plus efficaces, et contribuent à faire revenir volontairement des personnes qui, ensuite, peuvent témoigner que l'Europe n'est pas nécessairement la terre promise ? Attention aussi aux gouvernements qui vous donnent tous les laissez-passer consulaires que vous réclamez, mais ne font rien contre les réseaux de passeurs. Mieux vaut des partenaires rudes et fiers plutôt que ceux qui adaptent ce qu'ils vous disent à ce que vous voulez entendre et jouent sur les deux tableaux. Il faut enfin en finir avec la politique du chiffre, qui conduit à faire des réadmissions « Dublin », dont on sait parfaitement qu'elles n'éloignent la personne que pour quelques jours, ce qui ne change rien à la situation réelle. Tout cela se fait au mépris de la dignité des personnes concernées ! J'aimerais tant entendre

Nous en débattrons de nouveau dans quelques semaines, mais la réussite de cette politique passe par une plus grande harmonisation européenne, dans le respect total de nos principes et de nos engagements. Pour donner du sens à cette coopération européenne, il conviendrait de changer certaines attitudes. L'Europe ne peut pas être l'excuse de tous les échecs, alors qu'elle progresse chaque année sur la voie d'un système de plus en plus intégré de contrôle des frontières et de systèmes d'information interconnectés. Ainsi, à Roissy, en juillet dernier,

Ce n'est pas acceptable ! La progression de notre politique d'asile se fera en Europe et avec l'Europe. Madame la ministre, parce que votre politique n'est pas la bonne, le groupe socialiste et républicain refusera de voter ces crédits. La parole est à M. Stéphane Ravier. Madame

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, 3,6 milliards d'euros, c'est le budget de l'État pour réguler l'asile et lutter contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas rien ! Mais le plus intéressant, c'est non pas le montant de l'enveloppe, mais ce que vous en faites. la répartition, seulement 10 % vont à la lutte contre l'immigration clandestine, alors que la prise en charge des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande nous coûte 1,6 milliard d'euros, soit les deux tiers du budget de la mission. Si l'on considère que seulement 38 % des demandes d'asile sont acceptées, cela fait 1 milliard d'euros accordé à des personnes qui n'avaient pas le droit de venir en France. Ce milliard gaspillé aurait pu servir à expulser 77 000 clandestins, sachant que, parmi les 900 000 qui se trouvent sur notre territoire, 334 000 se sont manifestés pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État, qui leur est réservée, et dont le budget s'élève à 1 milliard d'euros, La réponse du Gouvernement ? La création de 6 000 nouvelles places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Les 100 000 Marseillais parqués dans des logements indignes, les 10 millions de Français qui survivent au-dessous du seuil de pauvreté et qui, pour nombre d'entre eux, n'arrivent plus à se soigner, apprécieront. Depuis des décennies, le nombre d'expulsions ne cesse de diminuer. Sur 65 000 mesures d'éloignement prononcées, à peine 10 % sont effectuées. À quoi sert la justice, mes chers collègues, si les décisions prises ne sont pas appliquées ? 1,2 million de titres de séjours ont été délivrés, soit les populations de Marseille et de Toulouse réunies. Vous battez un record en la matière, madame le ministre, avec 275 000 titres en 2019. Si ce n'est pas de la submersion migratoire, cela y ressemble fortement De grâce, épargnez-nous la réponse lacrymale sur le devoir d'accueil, ils sont seulement 13 % à venir pour raison humanitaire et seulement 15 % pour travailler. Les demandes pour motifs universitaires ou familiaux représentent 65 % du total. on le sait, l'immigration étudiante est une filière de l'immigration illégale. Le président Giscard d'Estaing avait d'ailleurs confessé l'erreur grave qui fut la sienne d'instaurer le regroupement familial, regroupement qui n'en finit jamais. Tant que vous n'inverserez pas les flux de l'immigration, notre pays continuera d'être submergé et sa population remplacée. Le budget doit être inversé : 90 % pour les expulsions et 10 % pour l'accueil. Avec cet argent, nous pourrions expulser l'ensemble des clandestins en seulement deux ans ! Elle est là, la chance de la France. Quant aux pays d'origine qui refusent d'accueillir leurs ressortissants, comme le Congo, la Bosnie, le Nigéria ou encore le Mali, la négociation devrait être simple vous avez besoin de notre argent, nous n'avons pas besoin de vos clandestins. Si vous voulez le premier, il vous faudra accepter les seconds. C'est simple, la politique, ... C'est simplissime ! ... y compris la politique migratoire, pour peu que l'on ait de la volonté. Votre volonté récente, madame la ministre, a été de fermer les frontières, mais pour empêcher les Français d'aller skier chez nos voisins, pendant que ces mêmes frontières restent totalement ouvertes à ce que le Président de la République défunt ». Cessez de faire parler les morts ! Il n'y a décidément que vous, madame la ministre, pour prendre des décisions aussi absurdes, et comme dirait M. Fernand de Montauban, l'équipe d'Emmanuel Macron, « elle ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît

On peut dire calmement, sans tout mélanger et sans agressivité, qu'avec près de 2 milliards

reconnaître un certain nombre de choses positives. Je tiens à noter une forte augmentation du budget, que ce soit en autorisations d'engagement ou en crédits de paiement, de l'action n° 03, Lutte contre l'immigration irrégulière, qui augmente de 15 % par rapport à 2020, 11, Actions d'intégration des primo-arrivants, en hausse de 9 % par rapport à 2020. Cela correspond aux objectifs fixés par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Hélas, ce budget ne permet pas de les atteindre. Les crédits de cette mission reposent sur les programmes 303, « Immigration et asile », et 104, « Intégration et accès à la nationalité française ». La mission « Plan de relance » complète les crédits de la mission à hauteur de 37 millions d'euros en autorisations d'engagement Le plan de relance prévoit effectivement le financement de 2 000 places complémentaires d'hébergement sous la forme de 500 places en centres d'accueil et d'examen des situations et de 1 500 places dans les dispositifs de préparation au retour favorisant l'éloignement aidé d'étrangers en situation irrégulière. Les rapporteurs pour avis de la commission des lois, Muriel Jourda et Philippe Bonnecarrère, ont indiqué que « les crédits de la mission s'inscrivent dans un contexte de pression migratoire toujours particulièrement intense », citant un nombre « record

toujours selon ce rapport, la pandémie pourrait anéantir vingt ans de progrès dans les luttes contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ce qui pourrait doubler le nombre annuel de décès.

De manière plus prosaïque, le programme 303, « Immigration et asile », comprend l'essentiel des crédits de la mission. Il vise à assurer le financement des politiques publiques relatives à l'entrée, la circulation, le séjour et le travail des étrangers, l'éloignement des personnes en situation irrégulière, ainsi que l'exercice du droit d'asile. À cet égard, l'action n° 02, Garantie de l'exercice du droit d'asile, constitue très nettement le premier poste budgétaire de la mission et finance les dépenses d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, l'allocation pour demandeurs d'asile et l'Ofpra. La forte croissance de la dotation accordée à l'Ofpra, notamment en 2020 et, dans une moindre mesure, en 2021 visait l'objectif d'une réduction des délais de traitement des demandes d'asile. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas permis de l'atteindre. Les délais risquent d'être Le programme 104 comprend quatre actions concourant à l'intégration des étrangers séjournant régulièrement en France, notamment ceux qui se sont vu reconnaître le bénéfice du droit d'asile. Après deux années de forte progression- 431 millions d'euros en 2020 -, ces montants se stabilisent à un niveau élevé. L'ambition du Gouvernement de renforcer sa politique d'intégration est bien réelle, mais les résultats peinent à être perçus, notamment en termes de maîtrise de la langue française, premier facteur d'intégration. Le contrat d'intégration républicaine n'a pas encore porté ses fruits. La crise sanitaire a eu un impact fort

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en matière migratoire, il y a urgence.

de 49 % par rapport à la moyenne du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ainsi, plus de 400 000 étrangers sont entrés légalement dans notre pays en 2019, et 3,5 millions y vivraient.

Cette ville souffre déjà assez. Pourtant, il existe des mesures simples, qui ont fait leurs preuves à l'étranger et que nous proposons depuis des années. Elles sont balayées d'un revers de main. la simplification du contentieux de l'éloignement, du durcissement des conditions du regroupement familial, des restrictions à la délivrance de visas aux ressortissants de pays non coopératifs qui ne délivrent pas de laissez-passer consulaires. Si le social n'a pas de prix, il a un coût.

Le système de prise en charge des MNA est au bord de l'implosion, faute d'une politique publique à la hauteur, et ce sont les plus vulnérables qui en sont les premières victimes. Sur le plan statistique, je rappelle que le ministère de la justice évalue à 20 000 le nombre de MNA, alors qu'ils sont en réalité 40 000.

Contrôlons plus strictement leur minorité ; généralisons le dispositif d'appui à l'évaluation de la minorité, le fichier AEM, qui a fait ses preuves. Et cessez d'abandonner les départements : il s'agit d'une compétence régalienne ! Permettez-moi d'insister une nouvelle fois sur la situation que nous subissons aujourd'hui dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

mes chers collègues, à voter contre ces crédits, qui sont très largement insuffisants au regard des enjeux et des souffrances vécues tant par les personnes en situation illégale que par les Français qui subissent toutes les décisions que prend

Madame le président, madame la ministre, mes chers collègues, qu'il me soit permis de rendre hommage à la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, qui a toujours plaidé pour l'unité des Français. Or cette dernière est plus que jamais menacée : la France est en guerre, non pas seulement contre un virus, mais bien contre l'islamisme radical, qui veut détruire notre nation et rejette toutes les valeurs qui fondent notre République et notre art de vivre. d'ailleurs, et fort heureusement, reconnu cet état de fait, nous continuons à débattre sur des évolutions budgétaires minimes sans nous donner les moyens de mener cette lutte avec efficacité et pragmatisme afin d'obtenir les résultats escomptés. Pourtant, indéniablement, les moyens sont là ; j'en veux pour preuve le déblocage, en quelques jours, de tous ces milliards d'euros pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, alors qu'on se contente de bricolage contre l'islamisme radical. : attaque au couteau rue Appert. L'auteur : un Pakistanais entré en France en 2018, demandeur d'asile. Vendredi 16 octobre : décapitation au couteau à Conflans. L'auteur : un Russe d'origine tchétchène, fils de réfugié politique. 29 octobre : meurtres au couteau dans la basilique de Nice. L'auteur : un réfugié tunisien arrivé à Lampedusa le 20 septembre. Certains crieront à l'acte isolé ou à la stigmatisation, et continueront à pratiquer la politique de l'excuse, préférant fermer les yeux, se boucher les oreilles ou se taire. Il y a urgence à regarder la réalité en face sur les conséquences de la crise migratoire, sans faux-semblants ni naïveté ; comme membres du Gouvernement ou du Parlement, notre responsabilité collective est engagée à l'égard des Français et au regard de l'histoire. « Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde ». Or une politique migratoire laxiste combinée à un droit d'asile inadapté et à une générosité dévoyée crée un appel d'air pour l'immigration illégale, qui est sur le point de nous submerger ; une partie de ces migrants, rejetant nos principes les plus fondamentaux, gangrène nos cités et remet en cause notre modèle républicain d'intégration, aujourd'hui en péril. Le problème n'est pas nouveau, mais il atteint un niveau de dangerosité inégalé. Les conditions créant ce terreau fertile sont connues et nous avons depuis trop d'années, sans doute, refusé d'en prendre la mesure,

d'abord, bloquer efficacement les frontières extérieures de l'Europe, cette Europe dont la fonction principale devrait être de protéger ses ressortissants vis-à-vis de l'extérieur avant de produire des normes qui les entravent à l'intérieur.

ensuite, fermer le robinet de l'immigration illégale et ne pas nous interdire de pratiquer une immigration choisie assumée. Une telle pratique n'est absolument pas contradictoire avec le respect du droit d'asile, auquel nous sommes toutes toutes et tous attachés. Il nous faut, enfin, refondre les règles d'acquisition de la nationalité française. Devenir Français est une chance, un honneur ; cela se mérite et ne peut être un simple droit automatique. Aujourd'hui prisonniers d'une législation trop permissive et trop tolérante à l'égard de ceux qui nous ont déclaré la guerre, nous devons nous réarmer, juridiquement et moralement. Nous n'avons pas à nous excuser d'être ce que nous sommes une grande nation, héritière de traditions millénaires aussi bien que de la pensée des Lumières, qui a foi en l'homme et est profondément généreuse à l'égard de ceux qui sont réellement persécutés dans leur pays. Mais cela n'implique pas de tout accepter sans mot dire et, surtout, de nous priver de nous défendre. Si nos institutions et les gouvernants n'agissent pas, demain ils feront face à la rue.

En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Béatrice Gosselin, dont le mandat de sénatrice commence le 4 décembre, à zéro heure.

aujourd'hui les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », qui sont, vous le savez, fortement mobilisés pour répondre à une politique migratoire que nous voulons maîtrisée et équilibrée. Cet équilibre repose, dans la droite ligne de la volonté du Président de la République depuis 2017, sur une politique d'humanité dans l'accueil et dans l'intégration, mais aussi de clarté à l'égard de celles et de ceux qui entrent irrégulièrement sur le territoire national ou qui s'y maintiennent, bien que déboutés de leur demande d'asile.

prévoit une augmentation des crédits de 36,8 millions d'euros, soit de 2 %, par rapport à la loi de finances initiale pour 2020. Et je concentrerai mon intervention sur la question budgétaire, qui nous réunit ce soir.

tout d'abord : les principales dépenses en matière d'asile, dans ce programme, portent sur l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile. Cela se traduit par une hausse significative du budget consacré à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)

Les actions menées en matière d'hébergement auront elles aussi un effet sur la dépense consacrée à l'ADA. À ces actions s'ajoutent des moyens financiers importants. Le point fort du PLF pour 2021 en matière d'hébergement, c'est la création de 6 000 places supplémentaires

L'amélioration des délais de traitement de la demande d'asile est une priorité de notre action en la matière, parce qu'elle doit nous permettre d'accueillir dignement celles et ceux qui ont droit à la protection de la France et,, de répondre rapidement à celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester durablement sur le territoire.

et ces 200 ETP supplémentaires sont déjà en poste, recrutés, formés, opérationnels. Mieux lutter contre l'immigration irrégulière, ensuite : le Président de la République, en déplacement le mois dernier dans la zone frontalière du Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, a annoncé un doublement des forces de sécurité déployées aux frontières. L'investissement immobilier concernant les centres de rétention administrative témoigne également de la volonté résolue du Gouvernement. Trop souvent, le manque de places en CRA a fait obstacle à l'éloignement ; 29,4 millions d'euros seront consacrés au financement de la tranche 2021 de ce plan d'extension des CRA.

d'euros. J'ai ainsi souhaité, par exemple, accélérer la naturalisation des travailleurs étrangers qui ont été en première ligne pendant le confinement. Nous avons d'ores et déjà reçu 1 419 demandes de la part des préfets. Parmi les autres actions, je tiens à citer celles qui concernent la maîtrise de la langue française, la formation civique pour le partage des valeurs de la République et la participation à la vie de la société, l'accès à l'emploi, la prise en charge de certaines situations particulières comme celle des réfugiés, et singulièrement des réfugiés yézidis, que le Président de la République s'est engagé à accueillir sur le sol français- je pense notamment à ces femmes et enfants yézidis qui ont survécu au génocide perpétré par Daech en Irak. Ces actions sont essentiellement portées par l'OFII, mais aussi par des porteurs de projets et des opérateurs dans les territoires. Pour ce qui est de l'OFII, les crédits d'intervention prévus pour 2021 s'élèvent à 11 millions d'euros.

aux crédits consacrés à l'accompagnement des réfugiés, ils restent mobilisés pour le financement des centres provisoires d'hébergement, à hauteur de 8 710 places.

en France, en matière d'éloignement, beaucoup plus mal qu'ailleurs. L'Allemagne éloigne à peu près 55 % de ceux qui sont déboutés du droit d'asile ; la moyenne européenne est de

Les entretiens approfondis qui sont menés par les auditeurs de l'OFII au début et à la fin du parcours d'intégration républicaine améliorent d'ailleurs l'orientation, notamment vers le service public de l'emploi. Il ne nous semble donc pas utile

En effet, malgré la volonté affichée par le Gouvernement d'améliorer le taux d'exécution des expulsions prononcées, les crédits de la mission ne traduisent pas une orientation budgétaire en ce sens. Les crédits de l'action n° 03, Lutte contre l'immigration irrégulière, sont en quasi-stagnation,

à 7,8 % pour les six premiers mois de 2020, en raison de l'épidémie de coronavirus. L'incapacité de la France à expulser les clandestins est particulièrement préoccupante ; elle nuit à l'intégration des immigrés en situation régulière, comme l'a d'ailleurs souligné la commissaire européenne en charge des affaires intérieures devant le Sénat le 5 novembre 2020. Comme le rappelle la Cour des comptes dans un rapport de mai 2020, l'échec de notre politique d'expulsion s'explique aussi par des raisons juridiques : non-délivrance des laissez-passer consulaires, difficultés d'identification des personnes concernées par les OQTF, souveraineté des États en matière d'autorisation d'atterrissage des avions, etc.- la liste est beaucoup trop longue. Le Gouvernement s'est engagé à travailler sur ces sujets des négociations avec les pays concernés. Ce thème a notamment été abordé à l'occasion de la tournée au Maghreb entreprise en novembre 2020 par le ministre de l'intérieur. Si ces négociations venaient à aboutir en 2021, les crédits destinés aux frais d'éloignement prévus dans le PLF pour 2021 seraient largement insuffisants pour financer la hausse des expulsions.

nous avons est un débat budgétaire, mais ces sujets ne sont en rien budgétaires. Notre collègue a tout à fait raison de dire que le taux d'éloignement

le problème n'est en rien budgétaire ; cela ne sert à rien, mes chers collègues, de consacrer 10 millions d'euros de plus à l'éloignement. Les problèmes que l'on rencontre sont d'une tout autre nature,

depuis 2014. Cet effroyable seuil a été franchi en mars 2020, le naufrage d'un bateau au large des côtes libyennes ayant entraîné la mort de 91 personnes migrantes. La Méditerranée se transforme en cimetière et, par son inaction, l'État français se fait complice de ces morts. Il est temps que cela cesse Nous nous devons de porter assistance à ces enfants, à ces femmes et à ces hommes naufragés. Arrachés à leur terre natale par les affres de la vie, les guerres ou l'instabilité politique, ils n'aspirent qu'à une chose trouver la paix en Europe, en attendant de pouvoir rentrer un jour dans leur pays d'origine. Ainsi est-il proposé de créer un programme intitulé « Sauvetage des naufragés des naufragés » qui financerait des dispositifs maritimes affrétés par l'État français afin de porter secours aux embarcations de fortune en détresse. Le financement de cette mesure se ferait un prélèvement de 12 millions d'euros, soit le double du budget de l'ONG SOS Méditerranée, sur les crédits de l'action n° 03, Lutte contre l'immigration irrégulière. La France, pays des droits de l'homme, se doit d'être à la pointe de la solidarité

dit de « répartition » des personnes qui sont débarquées après leur sauvetage en Méditerranée. Par exemple, à La Valette, le 23 septembre 2019, la France a obtenu un accord de l'Italie, de Malte et de l'Allemagne sur un texte visant à préciser les modalités de débarquement et les relocalisations qui s'ensuivent afin de pouvoir sauver autant que possible les personnes qui sont dans ces embarcations. Nous poursuivons cette action en vue d'une approche solidaire des États de première entrée dans le cadre du dialogue européen. Dès lors, le Gouvernement est défavorable à la

Je voudrais en profiter pour restaurer l'image de Marseille, qui a été un peu dégradée par les interventions de deux de mes collègues. Ils l'ont citée comme étant une ville submergée par l'immigration.

est faite au financement de la lutte contre l'immigration irrégulière, au détriment de l'intégration et de l'accès à la nationalité française. En effet, depuis 2017, les crédits accordés à la police aux frontières ainsi qu'aux actions de répression des personnes migrantes sont en augmentation constante et disproportionnée, à hauteur de 61,8 %. Obnubilé par sa chasse électorale à droite, le Gouvernement en oublie l'essentiel. Le financement du programme 104, « Intégration et accès à la nationalité française », connaît une augmentation extrêmement timorée de 0,4 % dans ce PLF pour 2021. Ce programme est pourtant essentiel puisqu'il vise à donner un accueil digne aux personnes migrantes et à assurer leur suivi sur notre territoire, notamment en matière d'intégration, d'apprentissage du français et d'insertion sur le marché du travail. Ces actions semblent néanmoins bien secondaires à l'exécutif, qui préfère se concentrer sur une politique visant à décourager les migrants de rejoindre notre sol alors même que ceux-ci fuient les guerres, les famines, l'instabilité politique et, parfois même, les dérèglements climatiques. Afin de doter la mission « Immigration, asile et intégration » d'un budget plus équilibré et plus humain, il est proposé, par le présent amendement, de prélever 10 millions d'euros alloués à l'action n° 03, Lutte contre l'immigration irrégulière,

dans son PLF pour 2020 d'augmenter de 20 millions d'euros le budget de fonctionnement de l'Office. Nous avions noté avec intérêt cette amélioration, certes insuffisante, mais qui constituait un progrès au regard des moyens alloués les années précédentes. Cet effort ne s'est malheureusement pas inscrit dans la durée, puisque, dans ce PLF pour 2021, l'augmentation des crédits accordés à l'action n° 02, Garantie de l'exercice du droit d'asile, a considérablement diminué. Madame la ministre, pourquoi ce ralentissement ? Au sein de l'Ofpra, certains dysfonctionnements sont encore à déplorer. Les services de l'Office sont engorgés et ne peuvent examiner correctement les dossiers des demandeurs d'asile dans des délais convenables. Cette réalité s'est d'ailleurs encore accentuée pendant la pandémie, puisque le temps de traitement moyen d'un dossier a été, cette année, de 241 jours, contre 161 jours en 2019. Cette situation est regrettable et requiert que davantage de moyens soient injectés dans le fonctionnement de l'Ofpra, afin que l'effort budgétaire enclenché l'année dernière se poursuive durablement. Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien à la garantie de l'exercice du droit d'asile à hauteur de 5 millions d'euros. Ces moyens viendraient appuyer le recrutement de personnels qualifiés, mais aussi la formation des agents des agents déjà en fonction afin qu'un traitement plus fluide des dossiers soit effectif au sein de l'Office. Quel

des interprètes, des ouvriers polyvalents, des cuisiniers, des physionomistes, soit environ 800 personnes sans lesquelles l'armée française aurait été sourde et muette en Afghanistan. Ces gens ont été absolument abandonnés à leur sort quand la France a quitté l'Afghanistan. Très peu d'entre eux ont pu avoir la possibilité de venir en France. En revanche, ils ont été, comme les harkis jadis, poursuivis par leurs concitoyens comme étant des traîtres, car ils avaient travaillé pour l'armée française. Le journaliste Quentin Müller a mené une enquête, pour ne pas dire une croisade. Aujourd'hui, certains interprètes de l'armée française et leur famille ont fini par arriver en France. Ils sont soutenus par des bénévoles

financement pour régler le problème de cette centaine d'interprètes de l'armée française. Madame la ministre, cette affaire est la honte de la France. On ne peut pas avoir utilisé des gens en Afghanistan dans des conditions pareilles et les abandonner absolument à leur triste sort, car ces personnes sont aujourd'hui victimes d'attentats. Beaucoup d'entre elles sont déjà mortes. Il faut absolument que la France puisse accueillir celles qui restent. Quel est l'avis de la commission ? Je comprends

en Afghanistan, près de 800 personnels civils de recrutement local, les PCRL, dont une majorité d'interprètes, vous avez raison, ont oeuvré au profit des forces françaises déployées en Afghanistan entre 2001 et 2014. Après le retrait effectif de nos troupes d'Afghanistan, le gouvernement français a mis en place un dispositif en faveur de ces personnels. Il prévoit une indemnisation forfaitaire pour leur permettre la relocalisation dans une autre région d'Afghanistan, dans un pays tiers, au choix, ou pour ceux faisant l'objet de menaces graves, une procédure de relocalisation en France ou dans un autre pays. La France a mis en place ce dispositif pour eux, pour leur famille élargie et comprenant les parents jusqu'aux deuxième et troisième degrés. La relocalisation s'est bien déroulée, et elle s'est faite en trois phases entre 2012 et 2019. Au terme de ces trois phases d'examen, je vous annonce que 768 personnes se sont vu délivrer des visas d'installation en France. À leur arrivée, 408 cartes de résident leur ont été délivrées, ainsi qu'aux membres adultes de leur famille. Lors des deux dernières phases, ces personnes ont bénéficié d'une prime d'aide à l'installation, d'un accompagnement social, de la mise à disposition de logements. Lors de la dernière phase, la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés a été chargée de leur prise en charge et a mandaté un opérateur particulier, France Horizon. L'ensemble de ce dispositif a permis à la France d'exprimer sa reconnaissance, mais aussi de respecter ses engagements humanitaires à l'égard de ces personnels.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à périmètre constant, le budget de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » augmente d'un peu plus de 200 millions d'euros pour financer les élections départementales et régionales. Vous le savez, un projet de loi relatif à leur organisation sera bientôt déposé au Parlement. Les élections devront vraisemblablement se dérouler en juin prochain, suivant en cela les recommandations du rapport de Jean-Louis Debré, remis au Premier ministre le 13 novembre dernier. À périmètre constant, le budget de la mission doit se stabiliser en 2021 : l'effort se réduit pour les administrations de la mission, tout particulièrement pour l'administration territoriale. Ce point me paraît essentiel : après plusieurs années de baisse des crédits et des emplois de l'administration d'État dans les territoires, l'année 2021 pourrait marquer, et il était temps, un coup d'arrêt. En 2021, la mission sera principalement marquée par la poursuite de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (OTE). Celle-ci a été enclenchée par la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, mais son déploiement a dû être ralenti en 2020 du fait de la crise sanitaire et économique. Au-delà des questions qu'elle peut susciter, cette réforme semble interrompre une logique gestionnaire, de rabot sur les moyens des services de l'État, entamée il y a une douzaine d'années par la révision générale des politiques publiques. La création des secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles, prévue initialement pour le premier semestre 2020, devrait être effective le 1 janvier prochain, de même que le transfert au ministère de l'éducation nationale des missions sport et jeunesse exercées par les directions départementales et régionales de la cohésion sociale. Si je conçois l'objectif d'optimisation du fonctionnement de l'administration territoriale de l'État, je considère qu'il y a lieu de s'interroger sur le calendrier retenu par le Gouvernement. En effet, la deuxième vague de l'épidémie de covid-19 mobilise fortement les services, qui doivent pouvoir parer au plus urgent et rester focalisés sur la gestion de crise. Maintenir un objectif de transformation à très court terme n'est pas pertinent, tant du point de vue de la bonne mise en oeuvre de la réforme que de celui de son acceptation par les services. généraux communs (SGC) a déjà dû être repoussée au-delà du premier semestre 2020, mais, la crise étant toujours aussi prégnante, la date du 1 janvier prochain ne me paraît pas en phase avec la situation actuelle. En effet, je considère que le calendrier doit être adapté à l'ambition affichée par le Gouvernement : si la réforme de l'OTE est véritablement structurante, comment expliquer qu'elle ne puisse être différée de quelques mois et doive impérativement se dérouler dans le contexte de crise sanitaire majeure que nous traversons ? À titre de comparaison, la réforme des services économiques de l'État en région a, quant à elle, été ajournée ! Par ailleurs, au-delà de la limitation de la pression sur le budget et les emplois de la mission, des interrogations demeurent sur l'évolution du rôle de l'État dans les territoires. Les thématiques portées par la mission sont nombreuses et je n'ai malheureusement pas le temps de les évoquer toutes ici. Le principal sujet concerne l'accessibilité des services publics et, de ce point de vue, je tiens à rappeler que, même plus accessible, le « tout numérique » n'est pas une solution : il est indispensable de maintenir un accompagnement physique des personnes. Je pense, en particulier, à la dématérialisation des demandes de titres, qui a laissé de côté les publics les plus fragiles,

Je souhaite enfin évoquer le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui couvre également des actions relatives à la radicalisation. Alors que le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation devrait voir son rôle renforcé l'intégration de nouvelles missions liées à la prévention des dérives sectaires et au « contre discours républicain », je tiens à relever que les crédits du FIPD devraient baisser. En effet, pour 2021, l'action consacrée au FIPD affiche une baisse de plus de 3,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 3,9 millions d'euros en crédits de paiement. Je propose donc un amendement de crédits sur le FIPD de 3,84 millions d'euros afin de porter ces montants au niveau que vous avez annoncé, madame la ministre, sur votre compte Twitter. La prévention de la délinquance et de la radicalisation ne peut en aucun cas constituer une variable d'ajustement budgétaire. Il faut conclure. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, j'émets certaines réserves à l'égard du budget qui nous est proposé. Cependant, alors que la logique de rabot semble être remise en cause ... Merci,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » n'appelle pas d'observations particulières en ce qui concerne le programme 232- la forte augmentation des crédits étant nécessaire au regard de l'actualité électorale de l'année 2021 -et le programme 216, dont le budget s'inscrit dans la continuité de l'année passée. En revanche, nous ne saurions nous satisfaire de la stagnation des moyens humains et financiers consacrés au programme 354, Administration territoriale de l'État », dont les crédits reculent de 3,7 % en autorisations d'engagement et augmentent très légèrement, de l'ordre de 1,7 % en crédits de paiement. Contrairement à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement en juillet dernier, la présence de l'État dans les territoires n'est pas renforcée par ce projet de loi de finances pour 2021. Pour la première fois depuis 2008, les effectifs du programme ne subissent pas de réduction, ce que nous saluons. Pour autant, cette stabilisation n'est pas suffisante pour répondre aux attentes des citoyens et des élus locaux, qui dénoncent depuis des années des réformes administratives incessantes et des réductions budgétaires drastiques. Ces dernières ont abouti à la suppression de 5 000 postes, soit 25 % des effectifs en douze ans, et ont fait de certaines sous-préfectures des « vaisseaux fantômes » de la République. Cette stagnation est d'autant plus regrettable que les objectifs fixés par le plan Préfectures nouvelle génération (PPNG), qui s'est achevé l'année dernière, ne sont toujours pas atteints en ce qui concerne le renforcement des effectifs des missions prioritaires 231 équivalents temps plein supplémentaires sont nécessaires pour remplir les engagements du PPNG, mais le projet de loi de finances pour 2021 ne prévoit aucune création de poste pour le programme 354, « Administration territoriale de l'État Nous ne pouvons donc nous satisfaire d'une telle situation à l'heure où nous traversons une crise sanitaire, économique et sociale majeure, qui nécessite un véritable renforcement de l'administration territoriale de l'État.

je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

de l'acte fondateur de notre démocratie : le financement des élections. Commençons par le programme 354. Au risque de me répéter, on apprend tout autant des priorités du Gouvernement en analysant les montants des crédits, leur évolution et leur ventilation qu'en étudiant les indicateurs de performance qu'il choisit. J'ai été étonné, par exemple, de voir le taux retenu pour l'indicateur sur le respect des visites de sécurité des immeubles de grande hauteur accueillant du public, révisé à la baisse, les moyens n'étant pas au rendez-vous pour combler et lisser la part des visites programmées en 2020 n'ayant pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. De là à dire que l'État cherche à faire des économies sur la sécurité ... Ce programme couvre également la délivrance de titres et prévoit d'ores et déjà, faute d'y mettre les moyens, un allongement d'un tiers des délais pour l'instruction des passeports biométriques et de plus de 50 % pour les cartes nationales d'identité électroniques, ces augmentations étant justifiées par l'anticipation de demandes accrues.

En ce qui concerne les attentes des collectivités envers l'État, le rôle des préfectures en matière de contrôle de la légalité, mais aussi de conseil, apparaît comme en légère diminution, ce qui peut sembler contradictoire à l'heure où devrait se développer le rôle de conseil de la représentation de l'État et où le couple préfet-maire serait le bon niveau de réflexion. Si la numérisation doit permettre une rationalisation des coûts, je profite de l'étude de ces crédits pour faire de nouveau part des inquiétudes émanant des élus de nos circonscriptions et du Défenseur des droits, qui voient les accueils physiques des services publics fermer les uns après les autres. La « start-up nation » est une belle ambition, mais les difficultés liées au numérique sont nombreuses. Le fossé n'est pas qu'entre les générations. La présence d'un interlocuteur permet souvent de sortir de situations kafkaïennes que l'administration a parfois le don de créer, mais aussi de résoudre : autant qu'elle soit joignable et accessible physiquement. Le programme 232 permet à chaque citoyen d'exercer pleinement son rôle, qu'il soit en position d'électeur ou de personne éligible. C'est aussi ce programme qui distribue le financement public aux partis politiques.

résolues. Je soulignerai, outre les écarts des coûts et la part variable de la propagande selon les élections, l'utilité environnementale limitée de l'impression de millions de professions de foi quand une part non négligeable des électeurs a accès à des informations d'autres moyens. Enfin, le programme 216 concerne la conduite et le pilotage des politiques du ministère de l'intérieur. Je relèverai l'annonce des nominations de « sous-préfets à la relance », créant une inquiétude quant à la multiplication des interlocuteurs. Le fonds interministériel de prévention de la délinquance est de nouveau en baisse sensible. Les actions de prévention sont remarquablement concernées par cette diminution : prévention de la radicalisation, prévention des violences faites aux femmes et aux familles, et prévention de la délinquance. La prévention et le financement d'actions de prévention en association avec les collectivités territoriales et le milieu associatif sont vraiment les parents pauvres de l'action du ministère de l'intérieur. Les crédits sont en baisse : la différence entre les besoins et les moyens serait risible si ce n'était pas si triste. Cela ne surprendra personne si, au vu des maigres montants inscrits sur la ligne budgétaire qui englobe l'aide aux victimes, l'aide en faveur des jeunes délinquants, mais aussi la sécurisation des sites sensibles aux risques terroristes, notre groupe propose une évolution importante de ces crédits. Il faut conclure. C'est pourquoi le groupe GEST ne votera pas ces crédits. La

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous débutons l'examen de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » dans un contexte où l'ordre républicain est menacé et où un engagement fort de l'État est attendu. Au sein de cette mission, pilotée par le ministère de l'intérieur, trois responsabilités fondamentales sont mises en oeuvre : garantir l'exercice des droits des citoyens dans le domaine des grandes libertés publiques assurer la présence et la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République ; mettre en oeuvre au plan local les politiques publiques nationales. Pour mettre en oeuvre ces responsabilités, les crédits de la mission sont en augmentation de 6 % par rapport à 2020, s'élevant ainsi à 4,2 milliards d'euros. Nous saluons cette augmentation, face à l'étendue de la tâche. Au travers du ministère de l'intérieur, c'est l'État dans sa proximité et son adaptation aux territoires qui s'exprime, et l'exercice des libertés individuelles et fondamentales des citoyens qui se manifeste. La mission se décline en trois programmes. Je m'attarderai quelques minutes sur le nouveau programme 354, « Administration territoriale de l'État ». Il porte les moyens du réseau préfectoral, mais également ceux des services placés sous l'autorité des préfets de région et des directions départementales interministérielles Pour 2021, le programme bénéficie de 2,37 milliards d'euros, soit 56,4 % des crédits de la mission. Il vise plusieurs objectifs. tout d'abord, du déploiement de la réforme de l'organisation territoriale de l'État, notamment par la mise en place des secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles, par une nouvelle étape de la modernisation du réseau des agents affectés au sein des services des préfectures et des sous-préfectures, en regroupant l'ensemble des ressources de préfectures, des DDI, voire des Le programme stabilise les effectifs des préfectures et sous-préfectures au niveau atteint en 2020. La transformation et la rénovation du réseau préfectoral entreprises par cette réforme sont à saluer. Les préfets et sous-préfets seront au coeur de l'action de l'État dans le cadre de la relance, et le couple maire-préfet démontre encore aujourd'hui toute sa pertinence. Le programme 354 mobilise également l'administration territoriale de l'État en faveur du développement du réseau France Services et assure, à l'horizon 2021, le déploiement d'une carte nationale d'identité électronique conforme aux standards européens. Ensuite, l'augmentation des crédits de la mission se justifie également par le programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative », en forte hausse du fait de l'organisation des futures élections, à hauteur de 437 millions d'euros en 2021,

finance des projets structurants du ministère de l'intérieur, bénéficiera de 33 % des crédits de la mission, soit 1,3 milliard d'euros pour 2021.

Je soulignerai également la situation du fonds interministériel de prévention de la délinquance, crédité de 65 millions d'euros pour 2021 répartis entre des programmes d'actions de prévention des violences faites aux femmes et aux familles, de prévention de sécurisation des sites sensibles au risque terroriste et de prévention de la radicalisation. Afin de mettre en oeuvre toutes ces actions, le groupe RDPI votera en faveur des crédits de la mission.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je le regrette, mais chaque année l'examen de cette mission nous conduit exactement au même constat, celui du recul de l'État dans nos territoires, notamment les plus ruraux. Ce recul, c'est l'effacement progressif des services publics de proximité au profit de la dématérialisation et du tout-numérique. Non pas que nous soyons opposés à ces progrès, mais ils se heurtent à plusieurs réalités pratiques. Tout d'abord, l'ensemble de nos concitoyens n'a tout simplement pas accès à une connexion internet haut débit suffisante.

On peut néanmoins noter que le Gouvernement est cohérent dans son objectif, puisque l'on constate une montée en puissance des crédits de la mission numérique au sein du programme 216, « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur des politiques de l'intérieur ». L'essentiel des 4,2 milliards d'euros des crédits de la mission sont concentrés sur le programme 354, « Administration territoriale de l'État ». Comme l'année dernière, l'augmentation des crédits de ce programme vient simplement acter l'augmentation du périmètre de la mission. concerne l'administration déconcentrée, on pourrait se réjouir que, pour la première fois depuis 2008, il n'y ait pas de baisses des effectifs. Hélas, la crise de la covid nous a ramenés à la réalité que je décrivais en préambule : celle d'une administration territoriale sous-dimensionnée. Je regrette, une fois de plus, qu'à cette réalité on réponde par moins d'État et moins de services publics. Nous pouvons également le constater au travers de la poursuite, malgré le contexte, de la restructuration du service des impôts sur nos territoires ruraux. Vous me direz que vous n'êtes pas responsables, et vous aurez raison : c'est le fruit des politiques menées depuis de nombreuses années. Qu'elles s'appellent « révision générale des politiques publiques » ou « modernisation de l'action publique », l'objectif est toujours le même : réaliser des économies,

force est de constater que les 30 équivalents temps plein prévus sont insuffisants par rapport à la demande en ingénierie dans nos territoires. Un autre exemple est celui des maisons de services au public, dites aussi France Services. Là encore, l'État prend trop peu sa part et les deux tiers des maisons créées sont financées par les collectivités. viens au programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative ». Comme l'année dernière, il connaîtra une hausse de ses crédits du fait de la tenue des élections régionales et départementales. À ce titre, et à la suite des recommandations de Jean-Louis Debré, il nous faudra voter pour le report en juin de ces élections, mais également prévoir les surcoûts que cela occasionnera. Enfin, la disparition de la mission couplée à la baisse du fonds interministériel de prévention de la délinquance, dans lequel elle a été fondue, nous inquiète quant à la priorité que le Gouvernement accorde à la lutte contre les dérives sectaires.

je commencerai par un mot sur la gestion de la prévention de la radicalisation. Comme chaque année,

sur le point suivant : lors de la demande de carte nationale d'identité en mairie, les usagers présentent un certificat de naissance. Ce certificat de naissance peut être vérifié par les agents de la mairie le logiciel Comedec,

pour sécuriser les actes d'état civil ? Il suffirait de compléter l'article 47 du code civil par l'alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'État établit une liste de pays pour lesquels la présomption de l'alinéa précédent ne s'applique pas. Ce décret détermine les pays concernés et les modalités d'admission des documents destinés à prouver l'identité de leurs ressortissants. » C'est un véritable sujet ! Il faut établir- c'est très important -un plan de sécurisation de l'identité auprès des organismes sociaux le développement des outils de biométrie.

Un programme du Fonds européen pour la sécurité intérieure (FSI), doté de 3,8 millions d'euros pour la période 2014-2020, va être reconduit. Peut-être est-ce le moment d'utiliser ces fonds européens

en légère augmentation par rapport à l'année précédente, soit +3,6 % en autorisations d'engagement et +6 % en crédits de paiement, il révèle, en réalité, une hausse en trompe-l'oeil en fonction des programmes budgétaire concernés. Cette mission appelle donc trois remarques. Tout d'abord, sur la présence de l'État dans nos territoires, avec le programme 354 : s'il est vrai que, pour la première fois depuis 2008, l'administration territoriale de l'État ne subit pas de diminution de ses effectifs en 2021, la stabilisation des moyens humains et financiers va à l'encontre de la déclaration de politique générale du Premier ministre du 16 juillet dernier. Or les préfectures, notamment de département, ont été progressivement dépouillées de leurs leviers d'action par les réformes menées depuis des décennies. Ainsi, dans de nombreux territoires, les moyens humains et matériels de l'État déconcentré sont aujourd'hui minimes, donc insuffisants, notamment- nous l'avons vu -pour faire face à la crise sanitaire, et ce malgré l'engagement des agents, que je tiens à saluer. Pour y répondre, le Gouvernement annonce la création d'une nouvelle catégorie de représentants de l'État, les sous-préfets à la relance. L'occasion est donc donnée de doter les services départementaux de l'État qui en ont le plus besoin de ces moyens exceptionnels. Or il n'y a rien de précis sur ce point dans le PLF, pas plus que dans les axes de déploiement de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. la territorialisation du plan de relance est la condition de sa réussite. Et seules les préfectures de département peuvent être l'échelle garante de l'efficacité escomptée. En outre, la nouvelle rationalisation proposée dans ce budget, associée à la montée en puissance de la direction numérique du programme 216, ne doit pas être synonyme, comme c'est trop souvent le cas, de baisse de la qualité de service, comme nous avons pu le constater avec la fermeture de trop nombreuses trésoreries locales. Ma deuxième remarque concerne les prochaines échéances électorales, dont le financement relève du programme 232. L'augmentation des crédits de ce programme explique, presque à elle seule, la hausse du budget de la mission. En effet, le calendrier de 2021 sera chargé, avec les élections départementales et régionales en mars prochain. Il faut donc anticiper certaines dépenses, notamment celles permettant de garantir la sécurité sanitaire. Mais il est regrettable que, malgré les leçons budgétaires que nous aurions pu tirer des élections municipales passées, l'éventuel report des élections au mois de juin et la majoration du plafond des dépenses de campagne, proposés par Jean-Louis Debré, ne soient pas budgétés dans le cadre de cet exercice budgétaire. ailleurs, madame la ministre, au nom des principes qui fondent notre démocratie, il y a urgence à lever le flou qui entoure la date des scrutins. L'absence de décision prend aujourd'hui en otages élus Ces rendez-vous sont des moments importants pour nos territoires et leurs habitants, qui ont besoin de lisibilité. Enfin, je souhaite faire part de mon incompréhension face à la baisse continue, depuis 2018, du budget alloué au fonds interministériel de prévention de la délinquance, alors que notre pays est confronté à une menace terroriste élevée, à une montée de la violence et à une radicalisation dont nous avons pu mesurer encore récemment les conséquences tragiques. et contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, cette mission a une incidence directe et très concrète pour nos compatriotes dans les territoires, surtout les plus ruraux. Le maillage territorial de l'État et sa capacité d'action dans nos territoires doivent être renforcés, à plus forte raison dans le contexte actuel, marqué par une crise sanitaire sans précédent, un ordre républicain abîmé et une société plus que jamais fracturée. doit prendre ses responsabilités et ne peut constamment se reposer sur les collectivités territoriales, pour lesquelles faire mieux avec moins n'est pas seulement un slogan, mais une réalité- fortement accentuée par le contexte financier de baisse attendue des recettes et d'explosion actuelle, mais aussi à venir, des dépenses. Je pense à cet égard aux conseils départementaux, à celui de l'Oise, que je connais bien pour avoir eu l'honneur de le présider, et qui va sûrement voir la charge du revenu de solidarité active (RSA) bondir, sans parler de celle relative aux mineurs étrangers isolés. Vous le savez, les collectivités agissent au coeur de la crise sanitaire pour préserver les services rendus à leurs administrés et pour limiter l'impact économique de ladite crise. En retour, elles doivent pouvoir compter sur l'État. Madame la ministre, constance et cohérence ont guidé mon intervention, par rapport à celle de l'année précédente.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'année 2020 est marquée par de nombreuses situations particulièrement difficiles auxquelles l'État doit fait face aux niveaux sanitaire, social, économique ou sécuritaire. Si ce contexte redéfinit nos priorités, il ne doit pas nous faire renoncer à maintenir et à renforcer l'organisation de l'État, bien au contraire ! Les épreuves que notre pays traverse actuellement nous montrent l'absolue nécessité d'assurer la continuité de l'action publique. Les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » que nous examinons ce soir soutiennent ce qui est au coeur de nos institutions républicaines. Cette mission revêt donc une importance primordiale, en visant trois objectifs : garantir aux citoyens l'exercice de leurs droits dans le domaine des libertés publiques assurer la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire ; mettre en oeuvre au niveau local les politiques publiques nationales. Les crédits de la mission prévus par la loi de finances pour 2021 s'élèvent à 4,2 milliards d'euros, en légère hausse par rapport à l'année précédente. Toutefois cette augmentation cache une évolution très disparate selon les programmes qui composent la mission. Ainsi, le programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative », dont les crédits financent l'exercice des droits des citoyens dans le domaine des élections, de la vie associative et de la liberté religieuse, enregistre une hausse particulièrement forte de ses crédits. Cette augmentation tient principalement à l'organisation des élections départementales et régionales, ainsi que des élections territoriales en Corse, en Martinique et en Guyane, prévues en 2021. Quant au programme 216, « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », auquel sont rattachés les moyens du pilotage des fonctions support, et de la gestion des affaires juridiques et contentieuses du ministère, il voit son budget croître très légèrement afin de permettre la poursuite des réformes engagées en 2020. Enfin, le programme 354, « Administration territoriale de l'État », qui supporte la majorité des crédits de la mission, comprend les moyens des préfectures, des sous-préfectures et des directions départementales interministérielles. Ce programme est fondamental pour les liens entre l'État, les collectivités et les citoyens. Après plusieurs années de coupes budgétaires drastiques, il voit ses crédits stagner, alors que le Premier ministre avait annoncé dans sa déclaration de politique générale, le 16 juillet dernier, que « les moyens de l'État [seraient] confortés dans leur action quotidienne ». Cette stagnation est particulièrement problématique à l'heure où, pour faire face à l'épidémie de covid-19, la présence de l'État dans les territoires aux côtés des citoyens et des élus locaux est plus que jamais nécessaire. Or, depuis quelque temps déjà, dans nos territoires ruraux, nous assistons à un recul des services publics, surtout des services de proximité. La dématérialisation et la mutualisation ont conduit à la suppression de nombreux points de contact qui permettaient à une population souvent âgée ou n'ayant pas accès à internet de disposer d'un interlocuteur dans ses démarches administratives. Si ce processus de dématérialisation est certainement nécessaire au vu des évolutions technologiques, il ne doit pas accroître la fracture numérique, territoriale et sociale. L'État doit entendre le sentiment d'abandon de nombreux habitants des territoires ruraux, entretenu par les suppressions successives des relais physiques de l'État dans leur commune au profit de services en ligne ou trop éloignés.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Administration générale et territoriale de l'État » est problématique cette année, à deux égards. D'une part, nous ne pouvons nous satisfaire que les crédits du programme « Administration territoriale de l'État » stagnent après plusieurs années de coupes budgétaires. Depuis 2008, ce sont 25 % des effectifs qui ont été supprimés. accuse ainsi un retrait au niveau local, retrait justifié par la rationalisation de la dépense publique, mais qui n'a abouti qu'à l'amoindrissement des services publics. Ce sont les moyens des préfectures et des directions départementales qui sont en jeu, ainsi que leur capacité à remplir des missions qui prennent d'autant plus d'ampleur depuis la crise. Le Gouvernement ne peut se contenter de parler du couple « préfet-maire », sans permettre à celui-ci de se développer, j'oserais même dire de « s'épanouir », sans risque de divorce Les élus locaux ont manifesté leur ras-le-bol depuis le début de l'examen de ce budget, face au manque de soutien financier et humain de l'État. Mais, depuis le début de la crise sanitaire, ils demandent aussi une amélioration de leurs relations avec l'État. Un soutien massif des services déconcentrés est impératif. À ce titre, la verticalité n'est pas une bonne méthode sans un minimum d'horizontalité, d'anticipation, d'échanges et d'accompagnement. Ce programme devrait être abondé en crédits pour améliorer le fonctionnement des services déconcentrés, d'autant plus que nous attendons pour 2021 la loi « 3D » ou « 4D », avec dans son titre au moins un « D » pour « déconcentration Mais on ne peut réformer l'organisation territoriale de l'État à moyens constants, alors que les collectivités ont besoin de renforcements concrets, constatables par les citoyennes et les citoyens. L'administration territoriale de l'État n'est pas en situation de faire face à la crise et aux sollicitations que rencontrent les élus quotidiennement. Pourtant, l'État s'appuie constamment sur les collectivités. Nous pensons par exemple aux maisons France Services, pour lesquelles l'État ne respecte pas aujourd'hui ses obligations d'affectation de deux emplois par maison. D'autre part, cette mission est importante cette année dans la mesure où son programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative », sera particulièrement mobilisé avec la tenue des élections départementales et régionales, d'où l'augmentation de 80 % des crédits. Mais il nous paraît compliqué d'évaluer les besoins, puisque nous sommes dans l'incertitude quant au calendrier électoral et aux conditions d'organisation de ces scrutins. Cette incertitude contribue notamment à maintenir une situation d'instabilité pour les élus locaux, qui ne peuvent assurer la relance des investissements publics dans ces conditions. Si le Parlement confirme le report des élections départementales et régionales au mois de juin 2021, le coût des mesures sanitaires qu'implique la mise en place de protocoles stricts conduira à une augmentation des crédits de cette mission. Nous devons nous assurer que tout sera fait pour que les conditions d'information des électeurs et d'égalité des candidats soient les meilleures possible. Le rapport remis par Jean-Louis Debré préconise en outre une majoration de 20 % du plafond des dépenses de campagne, qui n'est pas budgétée ici. Ce sont des enjeux démocratiques sur lesquels le Parlement doit avoir l'oeil, et la main. La tenue de ces élections ne peut reproduire le schéma du second tour des municipales. Le Parlement doit avoir la compétence exclusive pour décider d'un éventuel report. Pour toutes ces raisons, le groupe CRCE votera contre les crédits de

et donc de retrait de la présence de l'État dans les territoires, dans une logique de rationalisation de la dépense publique. La création des secrétariats généraux communs et la mutualisation des fonctions supports des directions départementales

Le programme reste stable, mais le financement est exogène, lié à la mission « Plan de relance » pour soutenir des projets numériques dont les enjeux sont très lourds.

Nous partageons les préoccupations de Mme la rapporteure spéciale sur les moyens du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). Ce programme doit garantir la continuité du service public et de la démocratie. La continuité du service public impose une action de proximité renforcée. Les réformes organisationnelles ne doivent pas se faire aux dépens de l'exercice de missions prioritaires, telles que le contrôle de légalité ou le soutien juridique aux collectivités.

ces points à plusieurs reprises. Il faudrait en réalité mobiliser le produit des économies réalisées pour renforcer l'accessibilité des services publics aux citoyens les plus fragiles et les plus éloignés du numérique.

la continuité démocratique, il est évident que parler d'une adaptation du calendrier électoral, en tant que telle, ne peut suffire.

la gestion des crises, la lutte contre la fraude documentaire, l'expertise juridique et le contrôle de légalité, ainsi que la coordination territoriale des politiques publiques. La dématérialisation intégrale des opérations de délivrance de titres réglementaires, lancée à la fin de l'année 2017, constitue une mesure phare

Le redéploiement de 1000 ETP vers les quatre missions prioritaires évoquées précédemment n'a pas été plus facile, en raison de l'absence de mobilité géographique, allant parfois à l'encontre de la rationalisation.

Force est de constater que le contrôle de légalité demeure encore perfectible, alors même que cette mission est garante d'une application uniforme de la règle de droit sur le territoire.

Heureusement, le dialogue en amont entre les élus et les préfets sur les sujets difficiles ou qui sortent de l'ordinaire permet d'aboutir à un faible taux de recours gracieux ou contentieux.

Cependant, comme j'avais eu l'occasion de le soulever lors des débats en séance publique, le rescrit ne saurait mettre les communes à l'abri d'un recours exercé par un particulier, un syndicat ou une association, et donc d'une éventuelle condamnation. Il serait intéressant de faire un bilan de cette mesure. Je terminerai en interrogeant Mme la ministre sur le sort réservé aux préconisations du rapport remis par le comité Action publique 2022. En réponse au constat d'une gestion en silo et d'une adaptation difficile des ressources aux enjeux prioritaires au niveau des préfectures, le comité préconisait de déconcentrer la gestion des ressources humaines et d'envisager la création d'une filière administrative territoriale interministérielle, en remplacement des corps administratifs actuels qui, gérés ministère par ministère, brident la mobilité. La création du programme 354, l'année dernière, répond à cette demande de mutualisation des moyens de l'État. La création, en 2021, de secrétariats généraux communs départementaux

et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle comprend les crédits de l'administration centrale du ministère, indispensables pour venir au soutien de l'activité opérationnelle de nos forces. De plus, elle abrite les crédits destinés au financement de la vie politique et à l'organisation des élections,

S'agissant de l'évolution des crédits par nature de dépense, je tiens à préciser que l'évolution des dépenses de personnels de la mission est marquée par l'absence de suppression d'emplois dans les préfectures et sous-préfectures.

Des réductions d'effectifs seront néanmoins réalisées sur les administrations centrales du ministère de l'intérieur ... Les crédits de masse salariale de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » progressent quant à eux de 21 millions d'euros, hors du compte d'affectation spéciale « Pensions

Nous avons souhaité que l'ensemble des personnels du ministère bénéficie d'un effort important en termes de conditions de travail, ce qui implique évidemment les effectifs relevant du secrétariat général et de l'administration territoriale. Ainsi, dans le périmètre de la mission, le parc automobile sera renouvelé par un effort supplémentaire d'environ 20 millions d'euros au titre de France Relance. Nous proposons également d'équiper les agents en doubles écrans et en informatique nomade pour favoriser le télétravail.

Je souhaite également dire un mot des grands projets numériques que nous menons et qui, nous semble-t-il, sont porteurs d'avenir. Il s'agit non pas de tout remplacer par le numérique, mais simplement de s'engager dans cette transition lorsqu'elle peut faciliter un certain nombre de dispositifs.

principalement en raison du fait qu'elle ne permet pas de garantir le caractère personnel du vote, au même titre que l'isoloir ou le déplacement des intéressés dans le cas de procurations. La proposition de loi déposée le 14 novembre dernier par l'auteur de cet amendement, notre collègue Éric Kerrouche,

Son budget a connu des baisses successives au fil des ans : en 2018, le fonds avait été très sérieusement amputé de ses moyens, enregistrant alors une baisse de près de 40 %.

Pourtant, ce fonds joue un rôle crucial pour la politique de prévention et les actions menées en faveur de la réinsertion de jeunes délinquants, ainsi que pour la prévention de la radicalisation et les actions de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Il permet enfin la sécurisation de sites sensibles au risque terroriste, tels que les lieux de cultes et les établissements scolaires. Nous sommes très surpris par la baisse de ce budget, qui nous semble en totale contradiction avec les engagements pris par le Gouvernement sur ces sujets.

et de la radicalisation, annoncée par Mme la ministre à l'issue du conseil des ministres du 27 septembre dernier.

ne l'aient pas été ! Heureusement, vous avez fait en sorte qu'il n'y ait pas de dégagement d'office, mais il y a tout de même un problème d'évaluation. À la même place que vous, une autre année, quasiment à la même heure, le ministre Bernard Cazeneuve s'était engagé à nous donner des évaluations que nous n'avons jamais obtenues. Certes, il y a un document de politique transversale, mais il nous faut des évaluations, madame la ministre.

Les contrats sont souvent de durée très courte- deux ou trois mois tout au plus -et s'enchaînent. Les contractuels sont gérés par les préfets qui peuvent être tentés de faire appel à cette ressource, même dans des cas où le recours à des agents titulaires serait justifié.

Nous proposons, pour l'ensemble de ces raisons, de renforcer les moyens du programme 354, « Administration territoriale de l'État », et son action n° 02, Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres. Quel est l'avis de la commission ? Si nous